j'ai le plaisir de saluer la présence, dans la tribune d'honneur, d'une délégation de trois parlementaires de l'Assemblée nationale du Koweït, conduite par M. Abdulkarim Al Kandari, président de la commission des affaires étrangères. La délégation est accueillie au Sénat par les membres du groupe d'amitié France-Pays du Golfe, présidé par notre collègue Jean-Marie Bockel. Elle se trouve en France dans le cadre d'une visite d'étude consacrée au renforcement des liens entre l'Assemblée nationale du Koweït et le Parlement français.

Cette visite fait suite à la mission menée au Koweït par une délégation du groupe d'amitié du Sénat en décembre dernier, qui a permis de souligner l'importance et l'intérêt des échanges entre nos parlements, ainsi qu'à une précédente mission koweïtienne, organisée en juin 2018. Le dynamisme de notre relation interparlementaire souligne aussi le rôle institutionnel du Parlement au Koweït. Il pourrait trouver une nouvelle expression dans des contacts prochains au niveau des présidents de nos deux assemblées, au Koweït ou en France.

L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Monsieur le président, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs,

Nous avons eu de longs débats, en commission spéciale puis en séance publique. Nous avons amélioré le texte ensemble, parce que, en tant que représentants des territoires, vous connaissez mieux que quiconque les besoins des entreprises. Vous savez qu'une entreprise ne se définit pas en premier lieu par sa taille ou son activité, mais par son territoire. Grâce à cette expertise, nous avons pu affiner le texte.

Pacte l'est en outre par les épargnants, auxquels la réforme de l'épargne retraite garantira plus de flexibilité, de liberté et de transparence. Attendu, Pacte l'est encore par les jeunes générations, car nous redéfinissons le rôle de l'entreprise dans la société en lui donnant la possibilité de se doter d'une raison d'être. Les jeunes générations attendent des entreprises qu'elles donnent un sens à l'économie, qu'elles se battent pour l'inclusion et pour une croissance durable : c'est ce que nous avons voulu affirmer en modifiant le code civil. Enfin, Pacte est attendu par notre industrie, car toutes ces mesures vont permettre de lever les blocages qui limitent la réindustrialisation de tous les territoires de France. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'en ai la conviction : la France fait face à des défis historiques, sûrement les plus brutaux et les plus décisifs des dernières décennies. les révolutions technologiques menacent de reléguer notre économie dans les dix prochaines années, non pas à la septième ou à la huitième place dans l'ordre des économies mondiales, mais à la dixième, voire à la quinzième, derrière le Mexique, le Brésil ou l'Indonésie.

Pacte répond à ces défis. Le rejeter, ce serait se résigner à ne pas les relever ; ce serait préférer abandonner notre souveraineté technologique, le combat pour une croissance durable et pour un capitalisme plus respectueux, plus égalitaire et plus conforme à notre tradition européenne ! La parole

a été dévoyé par les privatisations, qui auraient dû faire l'objet d'un projet de loi distinct. De fait, cette question, qui ne concerne nullement les entreprises, a masqué tout le reste, y compris dans les médias, au détriment même de la communication du Gouvernement envers les entreprises. En dehors des privatisations, ce texte aurait pu, et même aurait dû recueillir une large majorité dans les deux assemblées, autour de mesures utiles, à défaut d'être toujours ambitieuses ou novatrices. Des ouvertures étaient possibles sur de nombreuses dispositions, comme nous l'avons constaté en première lecture, mais peu ont été suivies d'effet, même si un certain nombre d'apports du Sénat- pas les plus importants -ont été conservés par l'Assemblée nationale. Nous avons le sentiment que ces ouvertures ont été victimes des privatisations, alors qu'elles prolongeaient la logique initiale du projet de loi, au service des entreprises. Sur la question des seuils d'effectifs, par exemple, nous avons relevé à cent l'ensemble des seuils aujourd'hui fixés à cinquante salariés dans le code du travail, un niveau qui constitue un réel frein à la création d'emplois et à la Nous étions prêts à trouver un compromis autour de soixante-dix, un seuil qui a du sens du point de vue économique, tout en excluant du dispositif les institutions représentatives du personnel. Nos collègues députés n'ont pas saisi cette occasion. S'agissant de la réforme du contrôle légal des comptes, je rappelle que nous en avons accepté l'économie générale, alors même que nous avions de sérieuses réserves quant à son incidence sur la sécurité financière des sociétés, sur la profession et sur le maillage territorial des petits cabinets. Outre des modalités de contrôle renforcées dans les groupes, nous avons proposé un report de l'entrée en vigueur de la réforme à 2021, pour permettre à la profession de s'adapter à ce changement brutal et de développer de nouveaux services. Sauf pour l'outre-mer, ces ajustements n'ont pas non plus été pris en compte, et la réforme s'appliquera dès le 1 septembre 2019. L'Assemblée nationale n'a pas davantage conservé le droit pour les actionnaires minoritaires d'obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes, même si elle a réintroduit cette faculté, sous une autre forme, me semble-t-il, dans la proposition de loi sénatoriale de simplification du droit des sociétés, examinée à la fin du mois de mars dernier et qui devrait revenir prochainement

Elle a rétabli l'obligation de conclure des conventions avec les régions pour la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. S'agissant du stage préalable à l'installation pour les artisans, l'Assemblée nationale a supprimé de nouveau purement et simplement toute obligation, alors que le Sénat avait proposé, dans une démarche de compromis, d'assouplir les modalités actuelles du stage, tout en lui conservant un caractère obligatoire. À l'instar de notre commission spéciale, qui n'a pas été suivie en séance publique, l'Assemblée nationale a aussi fait le choix de maintenir la faculté pour l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, de s'opposer à la délivrance d'un brevet dépourvu d'activité inventive ou d'application industrielle. veiller, madame la secrétaire d'État, aux moyens humains de l'INPI, pour que celui-ci puisse assurer de manière effective cette nouvelle mission. Pour ce qui est de l'interdiction des produits en plastique à usage unique et des produits phytopharmaceutiques, l'intervention du Sénat a été utile, en permettant de revenir sur les excès de textes récents. Nos collègues députés ont globalement suivi nos propositions sur le fond, ce dont il faut se féliciter. Enfin, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a renoncé à la création d'une nouvelle délégation parlementaire à la sécurité économique, votée en première lecture sans aucune concertation avec le Sénat.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici de nouveau réunis pour débattre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Comme, manifestement, c'est la dernière fois, je tiens, au nom du groupe Les Indépendants, à saluer de nouveau le travail de la commission spéciale et de ses trois rapporteurs, Élisabeth Lamure, Michel Canevet et Jean-François Husson, sous la présidence de Catherine Fournier.

Par principe, comme l'orateur précédent, je le regrette, parce que je pense que le débat est toujours utile en soi, même quand on craint de ne pas avoir le dernier mot.

motion. En effet, notre rôle, en tant que sénateurs, est de porter la voix des territoires dans le débat public. Très bien ! Quelle que soit l'issue du vote, je rappelle que ce projet de loi, globalement, va dans le bon sens : il apporte des solutions concrètes pour le développement de nos PME il encourage la création d'entreprises ; il soutient l'innovation et facilite une répartition plus équitable des richesses. Ce texte passe au crible toute une série de scories de notre droit : des blocages qui découragent la création d'entreprises, des carcans superflus qui brident l'innovation, des règles absurdes qui absorbent l'énergie de nos entrepreneurs. De ce point de vue, sincèrement, le projet de loi Pacte constitue une bonne nouvelle pour nos entreprises. Nos entrepreneurs étaient demandeurs.

Le Parlement a considérablement enrichi le projet de loi initial, malgré le contexte de la procédure accélérée, qui nuit à la qualité de notre travail. Le Sénat, notamment, a veillé à faire entendre la voix des territoires, avec un objectif clair : que les mesures ne restent pas hors-sol, mais répondent concrètement aux besoins des PME et ETI qui structurent notre tissu économique. Je pense tout particulièrement à l'amendement, déposé par notre groupe et adopté en première lecture, portant sur l'organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. L'Assemblée nationale, sur ce point, a entendu la voix du Sénat et gardé l'essentiel de nos dispositions. Nous maintiendrons ainsi dans nos territoires un réseau dense pour accompagner les entrepreneurs de proximité. Le Sénat a également soutenu des propositions ambitieuses que l'Assemblée nationale n'a pas conservées,

Sur ce texte comme sur tant d'autres, le Sénat s'est montré en même temps raisonnable et ambitieux. Raisonnable, car il a veillé, à l'heure où notre société paraît plus fracturée que jamais, à ce que tous les territoires bénéficient des fruits de la croissance. Ambitieux, car il a proposé d'aller encore plus loin sur nombre de mesures visant à libérer les énergies et à susciter chez nos concitoyens l'envie d'entreprendre. C'est pourquoi je regrette que les discussions aient achoppé sur les privatisations, tout particulièrement sur celle d'ADP. Le refus opposé à cette mesure, qui n'était pas dénué d'arrière-pensées politiques, nous a privés de l'occasion de nous faire entendre. Nous pouvions pourtant y apporter les garde-fous que nous jugions essentiels pour assurer à la puissance publique la pleine maîtrise du cadre dans lequel cette concession va s'opérer- car, mes chers collègues, elle va s'opérer. Je ne puis pas m'empêcher de penser que, si le Sénat avait suivi les recommandations de la commission spéciale, sa voix aurait davantage pesé dans la prise de décisions, et certaines des garanties intégrées en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale l'auraient été dès la première lecture au Sénat.

Les amendements proposés par la commission spéciale auraient permis de limiter les risques juridiques pour nos entreprises, tout en conservant la déclaration de principes. Le Sénat a opté pour la suppression pure et simple de l'article 61. Résultat : il a été rétabli dans sa rédaction d'origine, sans les garanties que nous espérions. Mes chers collègues, n'oublions pas la situation dans laquelle se trouve notre pays : il étouffe sous la pression fiscale et l'excès des réglementations Tout ce qui simplifie l'activité de nos entreprises et recentre l'État sur ses missions régaliennes redonnera du souffle à notre économie. Il y va de notre capacité à maîtriser notre destin dans un monde incertain. Il y va de notre capacité à maintenir une souveraineté nationale. nationale. Non, le débat n'est pas clos, tant s'en faut. Le Sénat a toujours des arguments à faire valoir et des positions à défendre, sur des textes qui ne sont jamais définitifs, quand bien même nous craindrions de ne pas avoir le dernier mot. C'est pourquoi

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

Elles sont impatientes de faire vivre la loi Pacte. Je ne doute pas qu'une large majorité de notre hémicycle soit intimement convaincue que cette loi est une bonne loi. Et pour cause : entre autres elle améliorera la parité femmes-hommes dans les directions des entreprises et créera un label pour les entreprises qui mènent une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées ; elle facilitera la création d'entreprises et réduira son coût ; elle simplifiera la croissance des entreprises en améliorant et diversifiant leur financement ; elle protégera leurs inventions et expérimentations ; elle financera l'innovation de rupture et protégera les entreprises stratégiques françaises. Je ne m'attarderai pas sur la partie tendant à faire évoluer le capital des entreprises publiques, mon collègue Richard Yung vous en parlera beaucoup mieux que moi. Je ne doute pas un instant, cependant, qu'il profitera de son temps de parole pour dénoncer la posture adoptée par certains

Je ne vais pas détailler toutes les dispositions qui composent ce texte, mais il est indispensable de revenir sur le projet audacieux que porte le chapitre III, symbole de liberté et de protection. Celui-ci réconcilie en effet performance économique et responsabilité sociale des entreprises. Il supprime le forfait social versé au titre de l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur l'ensemble des versements d'épargne salariale pour celles qui comptent moins il gèle l'intéressement au-delà d'un plafond, permettant ainsi d'améliorer son rendement pour les bénéficiaires ; il développe l'épargne salariale, ainsi que l'actionnariat salarié, et donne naissance à la société à mission

La notion d'intérêt social de l'entreprise et la nécessité de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux seront ainsi inscrites dans la loi par la modification de l'article 1833 du code civil. il instaure le fonds de pérennité, grâce auquel la France se dote d'un statut permettant de protéger de manière durable le capital de nos entreprises pour assurer leur croissance à long terme En réunissant tous ces éléments, ce chapitre donne un nouveau souffle aux entreprises, ce qui leur permettra d'innover, de créer et de se développer. Plus largement, de loi relève le défi majeur de la croissance des entreprises à chaque phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Pour cela, il transforme le modèle d'entreprise français, qu'il est temps d'adapter aux réalités du XXI siècle. pourtant être nombreux à estimer que les conditions ne sont pas réunies pour que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale soit adopté conforme, et à déplorer que cette dernière soit revenue sur un trop grand nombre de dispositions introduites par le Sénat. la raison d'être de la navette parlementaire et du bicamérisme ! N'oublions pas que l'Assemblée nationale a tenu compte de certaines améliorations apportées par le Sénat : quelque 99 articles ont été votés conformes, dont 13 articles additionnels issus de nos travaux. à la limitation des seuils d'effectif pour certains dispositifs fiscaux, à la possibilité, pour les majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, d'ouvrir un plan d'épargne en actions, un PEA, à la réforme de l'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale,

j'insiste sur le bon fonctionnement du bicamérisme, en vous rappelant que les deux chambres sont tombées d'accord sur nombre de suppressions d'articles. Certes, nos homologues ont enlevé des dispositions que vous aviez intégrées.

ou l'écart salarial d'un à vingt, suggéré par la confédération européenne des syndicats et que nous avions tenté d'inscrire en première lecture. C'est l'outil permettant de lutter contre l'écart incompréhensible des salaires que l'on observe dans certaines entreprises,

La rémunération est un facteur de bon fonctionnement de l'ascenseur social. C'est pourquoi cette mesure est si importante. Nous devons retrouver des critères de cohésion qui tirent l'ensemble des salariés vers le haut. En conclusion, c'est du mouvement que naît la croissance, et non de l'immobilisme. L'heure est venue pour la France de s'engager fermement dans cette voie. Le projet de loi Pacte en est un vecteur essentiel,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous restons clairement opposés à ce texte du Gouvernement, qui casse les seuils sociaux, détricote la Caisse des dépôts et consignations, supprime le stage préalable à l'installation des artisans et le recours aux experts-comptables. Alors que vous prônez la, vous brisez l'accompagnement à la création d'entreprises, avec pour conséquence l'échec du plus grand nombre. Pis, vous n'avez pas voulu légiférer sur le statut d'auto-entrepreneur, laissant les grandes plateformes numériques continuer à exploiter nos jeunes. Vous avez réformé l'épargne retraite, alors que vous vous apprêtez, pour répondre à la crise sociale, à allonger la durée de cotisation, à reculer l'âge de départ à la retraite et à casser la retraite par répartition. Madame la secrétaire d'État, nous n'avons pas dû visiter les mêmes ronds-points ou discuter avec les mêmes personnes, car je n'ai vu quant à moi aucune pancarte affirmant « Nous voulons mourir au travail ! Enfin, vous réalisez le tour de force de parler de partage de la valeur sans évoquer les salaires et leur augmentation. En 200 articles, ce qui devait être un pacte entre l'entreprise et l'État se transforme en pacte des loups entre l'État et les rapaces de la finance. Encore une fois, vous cédez aux revendications du Medef, offrant un panel de droits nouveaux au patronat, mais aucun pour les salariés.

et environnementale. Dans ces conditions, notre groupe ne prendra pas part au vote sur la question préalable. Alors que notre pays aspire à plus de justice fiscale et sociale, exige plus de citoyenneté et de démocratie sociale, vous répondez « compétition, libéralisme, profit. » Nous ne choisirons donc ni le parti de la droite sénatoriale ni celui de la droite gouvernementale. Pour nous, c'est blanc bonnet et bonnet blanc

Sans révéler ce qu'il contient- clause de confidentialité oblige -, je puis évoquer ce qu'il ne contient pas. On n'y trouve, par exemple, aucun recensement des 8 600 hectares que détient ADP,

Sans cela, comment fixer un prix ? Le bon prix est-il 10 milliards d'euros, quand 8 600 hectares en Île-de-France constituent une pépite inestimable, qui intéressera certainement bon nombre de promoteurs ?

qui sont rentables, et non les pistes elles-mêmes. Toutefois, s'il n'y avait pas de pistes pour que les avions décollent et atterrissent, il n'y aurait ni compagnies aériennes versant une taxe ni passagers qui consomment dans les magasins ! Il s'agit donc d'un raisonnement par l'absurde : peut-on dissocier l'autoroute du péage, la gare de la ligne de chemin de fer,

Loin de moi l'idée de vouloir répandre des, d'adhérer à une théorie du complot ou de relayer un « Vinci », mais souhaitez-vous toujours vendre l'ensemble des parts à Vinci,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle lecture de ce projet de loi fourre-tout comportant un ensemble de mesures qui n'ont souvent rien à voir les unes avec les autres.

Vous allez perdre chaque année 600 millions d'euros, qui ne reviendront plus dans les caisses de l'État. Où est le bon sens économique dans tout cela ?

de Toulouse et des autoroutes ont été des erreurs ? Nous poursuivons dans les mêmes travers ! Vous connaissez l'adage :

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à ce stade de l'examen du projet de loi Pacte, on ne peut exprimer que des regrets, voire une certaine frustration. En effet, l'échec de la commission mixte paritaire, suivi, vraisemblablement, du vote par le Sénat d'une motion tendant à opposer la question préalable, interrompt le dialogue entre les deux chambres et le Gouvernement, dans un domaine où une issue consensuelle ne me semblait pas hors de portée. Je vous avais fait part, en première lecture, de mes craintes concernant le périmètre de ce projet de loi, lequel contenait à mon sens des dispositions trop disparates, au détriment de sa cohésion. Qu'y a-t-il de commun entre la suppression du stage à l'installation des artisans, la possibilité de définir la raison d'être d'une entreprise et la privatisation de trois grands groupes publics ? Le résultat donne raison au dicton : qui trop embrasse mal étreint. Dans cet ensemble, on trouvait un gros caillou nommé Aéroports de Paris, sur lequel est venu se briser tout espoir de consensus.

totalement persuadé, car on pouvait évaluer différemment son opportunité financière en termes de dividendes hier et de revenus financiers demain. Il ne s'agit en aucun cas d'une opération de retrait patrimonial définitif,

les orientations générales de ce texte, destinées à favoriser la création et le développement des entreprises, en associant mieux les salariés à cette démarche. On peut ainsi saluer la simplification des procédures de création, de transmission et de reprise des entreprises, la rationalisation du nombre de seuils d'emplois et, surtout, l'introduction de souplesse lors de leur franchissement, le relèvement du seuil de certification des comptes, la suppression du forfait social sur l'intéressement pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et sur la participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés des aménagements pertinents concernant l'épargne retraite et l'assurance vie et la promotion d'un PEA-PME. Il ne s'agit là que de quelques exemples, qui viennent s'ajouter aux multiples dispositions de réduction de délais, d'allégement de contraintes et de simplification contenues dans ce texte. On peut cependant s'interroger sur certaines évolutions qui me semblent relever d'un affichage de simplification ou de modernité, dont l'impact à terme pourrait être incertain, voire négatif, pour les entreprises comme pour les territoires. La centralisation à l'échelon régional des réseaux consulaires est ainsi conforme à une évolution subie depuis quelques années, mais elle sera de nature à appauvrir les territoires éloignés des métropoles et des capitales régionales.

en matière d'accès au crédit et aux marchés pour les PME. En effet, à l'exception de dispositions concernant la gouvernance de la Caisse des dépôts et du groupe La Poste, le secteur bancaire semble avoir été laissé en dehors du texte,

s'agissant du souhait de faire de l'intéressement un marqueur du partage de la richesse produite par les entreprises en rendant ce dispositif obligatoire pour toutes les entreprises de plus de dix salariés. Cela répondait à l'objectif que se sont fixé le Gouvernement et le Président de la République, objectif qui ne pourra pas être atteint par de seules mesures incitatives. Dans les entreprises où ce dispositif déjà en vigueur, les salariés verront leur intéressement augmenter, car un dirigeant d'entreprise raisonne en enveloppe globale incluant la somme allouée et les taxes afférentes.

Dans le contexte actuel, cette mesure de justice sociale avait le mérite d'introduire du pouvoir d'achat, de valoriser le travail et de faire bénéficier l'entreprise de la motivation et de l'implication de ses salariés.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues,

Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises doit permettre aux entreprises françaises d'innover, de se transformer et de créer des emplois. Comment ne pas en partager les ambitions ?

texte, que le Gouvernement aurait pu soutenir s'il l'avait souhaité. Force est de constater que les députés sont largement revenus à leur rédaction de première lecture sur les principales mesures du texte. Les points d'accroche les plus symboliques sont connus l'évolution du stage préalable à l'installation des artisans, le doublement du seuil de cinquante à cent salariés, le refus d'un report à 2021 de la réforme du contrôle légal des comptes sans en modifier l'équilibre global, le rétablissement de la faculté, pour l'Institut national de la propriété industrielle, de s'opposer à la délivrance d'un brevet dépourvue d'activité inventive. En ce qui concerne la Française des jeux, les députés ont réinstauré la privatisation, tout en améliorant légèrement la régulation du secteur.

pour ceux qui sont à deux ou trois heures de l'aéroport. Mais, pour le reste, nous sommes en compétition avec les plus grands du monde. Ensuite, il faut poser la question en se rappelant que le capital de cette entreprise a été ouvert en 2006- c'est la droite qui en est

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, un « plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises », avouons que l'intention de ce texte était parfaitement louable et partageable. Mais c'était sans compter la fâcheuse habitude prise par le Gouvernement de tenter d'expédier, dans un flot de mesures d'ampleur et de nature sensiblement différentes, des sujets concrets et délicats. En l'espèce, le résultat ne s'est pas fait attendre. Ce qui devait être une loi sur un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises s'est piteusement transformé en loi sur la privatisation d'Aéroports de Paris Il aura fallu là encore, et par-delà la diversité des sensibilités politiques qui s'y expriment, que la quasi-unanimité du Sénat éveille les consciences en première lecture pour que le débat prenne enfin corps et que cette hasardeuse privatisation soit repoussée. Malheureusement bien sûr, par la suite, l'Assemblée nationale a réintroduit dans le texte les éléments favorables à cette funeste privatisation. Mais cela ne s'est tout de même pas fait sans mal

Je ne puis m'empêcher de relever, au passage, que, visiblement, le fameux non-cumul des mandats n'a pas amélioré l'assiduité en séance publique de nos collègues du nouveau monde La vérité, c'est que ce projet est, à juste titre, extrêmement contesté. À l'instar des échanges dont notre hémicycle a été le témoin lors de l'examen du projet de loi Pacte en première lecture, nos collègues députés ont réitéré leurs critiques sur « la mauvaise affaire », « la faute économique, stratégique et historique », l'erreur irréparable », synonyme d'un « abandon de souveraineté nationale » ; d'aucuns ont même mis en avant « un choix stupide », « un sacrilège Sentant le vent de la fronde monter au sein même du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, le 13 mars dernier, le Premier ministre s'est évertué à dépeindre Aéroports de Paris comme une entreprise fragile, mal gérée, dont l'État serait un actionnaire défaillant et qu'il faudrait donc mieux s'en séparer. Vous l'avouerez, c'est un argumentaire commercial surprenant pour qui cherche à vendre au meilleur prix Parallèlement, M. le ministre de l'économie et des finances a tenté de démonter, un par un, les arguments avancés- on peut d'ailleurs lui reconnaître une certaine constance en la matière. Il s'agirait non pas d'une privatisation, mais d'une simple concession pour soixante-dix ans- excusez du peu ! L'État stratège n'aurait pas vocation à diriger une entreprise concurrentielle. Il ne s'agirait pas de la privatisation d'un monopole. Ce n'est, certes, qu'un monopole régional, comme l'affirme justement le Conseil d'État, sauf que 80 % des visiteurs étrangers transitent en France par les aéroports parisiens ! Le sommet dans cette affaire, comme si cela ne suffisait pas, c'est l'indigence du cahier des charges de cinquante-six pages mis à notre disposition avec condescendance et consultable sur place, salle A 387, au troisième étage de l'aile ouest, au bout du couloir à gauche, exclusivement sur rendez-vous et aux heures d'ouverture s'il vous plaît ... des fois que l'on dérange ! Excellent ! Très bien ! La richesse de notre si belle langue française, le foisonnement des éléments de langage produits par Bercy ne sauraient nous faire prendre des vessies pour des lanternes, madame la secrétaire Cette opération est un mauvais coup pour la France. Cette opération est un mauvais coup pour les Français, qu'ils portent un gilet jaune ou pas ! Madame la secrétaire comme pour les autoroutes en leur temps, le Gouvernement aura bientôt à répondre de ce mauvais coup porté à notre pays, au moment même où il traverse l'une des crises les plus graves de son histoire récente. Enfin, pour quitter un peu le sujet Aéroports de Paris et conclure mon propos, à la suite du débat engagé autour d'une des mesures qui se voulait une mesure phare de la loi Pacte concernant le volet transformation des entreprises,

Au niveau de la foule immense que voilà, on éprouve comme une révélation. « " Je ne sais pas, disait, jadis, Louis Veuillot, quel souffle planant sur la multitude lui révèle qu'elle est une nation ". Nous tous, ici, en nous voyant nous-mêmes, nous connaissons que nous sommes un grand peuple qui s'assemble pour son salut. « Ce qu'il faut, c'est abolir l'humiliante condition dans laquelle l'organisation économique dérivée tient la plupart des travailleurs. Ce qu'il faut, c'est faire cesser le système en vertu duquel les intérêts de ceux qui apportent à la production leur travail s'opposent à ceux qui y apportent soit leurs biens, soit leur autorité, et qui fait que, dans une entreprise, les ouvriers sont des instruments et non pas des participants. Ce qu'il faut créer et faire vivre, c'est l'association du travail, du capital et de la direction qui confère à chacun la dignité d'un sociétaire responsable et bénéficiaire du rendement collectif pour sa part et à son échelon. Naturellement, on ne fera pas ça si on ne passe pas outre au sectarisme des spécialistes de la lutte des classes et, en même temps, aux routines de certains dirigeants et de certains capitalistes qui voudraient voir les affaires marcher toujours comme au temps de papa.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs,

d'autant qu'il ne tient pas compte, comme cela a été souligné par un certain nombre de mes collègues, de l'indemnisation éventuelle. En réalité, il n'y a aucune transparence sur ce projet du Gouvernement.

améliorer la situation dans les entreprises, lorsque l'on parle de la raison sociale. de la réserve foncière de 7 000 hectares dans le coeur de l'agglomération parisienne ? C'est le flou le plus absolu. le projet d'entreprise, nous avons du mal à comprendre s'il s'agit d'une entreprise bien gérée par la puissance publique, ou mal gérée, comme cela a été démontré par mon collègue, qui a cité les propos du Premier ministre.

des parkings des municipalités, 50 % des autoroutes, le CGD Express, la seule liaison de TGV concédée, et plusieurs aéroports sur le territoire national ? En réalité, il s'agit non pas d'une mise en concurrence- cela n'a rien à voir avec le libéralisme -, mais de la cession des bénéfices d'un monopole à une seule entreprise. L'environnement de la plateforme aéroportuaire, lui, n'est pas assumé financièrement. On le sait, il faudra sans doute doubler le trafic autoroutier, améliorer les liaisons ferroviaires avec la capitale et réaliser d'importants aménagements urbains. Mais là, les collectivités territoriales sont évidemment assez peu associées.

en ces termes : « Il nous paraît inconcevable que la privatisation puisse se faire au cours actuel ; la valeur économique de l'entreprise est largement supérieure. » Je crois que tout est dit cher collègue ! Compte tenu de la faible teneur des propos du Gouvernement, je me rallierai probablement à la motion référendaire, pour obliger l'État à écouter les citoyens.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, le titre était alléchant Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. » Il sonne comme un magnifique slogan publicitaire, sans en tenir, tant s'en faut, les promesses. Bâti sur les propositions du rapport Notat-Senard, il n'en retient qu'une dose homéopathique, espérant peut-être que le résultat final conservera la mémoire de la molécule première. En réalité, ce projet traduit un libéralisme exacerbé avec des effets toxiques pour les salariés, qui assurent la prospérité et la création de richesses. libéralisme dogmatique jusqu'à la caricature, mêlant dans un même élan les privatisations, la quasi-suppression des certifications, le refus d'un partage équitable de la richesse et le rejet d'une juste représentation des salariés dans les instances de gouvernance. des privatisations que rien ne vient justifier et dont on peine à saisir les véritables motivations, tant les explications sont laborieuses, les artifices si alambiqués que leur auteur, lui-même, semble ne pas y croire. Martial Bourquin a développé avec la force de conviction que je lui connais l'ineptie que représentent ces privatisations. Bernard Lalande et de nombreux sénateurs de tous horizons se sont émus du relèvement, sans ménagement ni délai,

et les seuils d'audit légal sont différents selon les pays qui ont bien intégré que « la confiance n'exclut pas le contrôle », en adaptant les seuils à la dimension de leur tissu économique et à sa territorialité. Deuxièmement, en supprimant le commissaire aux comptes dans les holdings en cascade, qui peuvent créer de nombreuses filiales dispensées de produire des comptes certifiés, vous donnez rendez-vous à l'opacité fiscale, à l'opacité sociale, à l'opacité financière, et ce malgré les recommandations du rapport Cambourg, qui vous appelait à sécuriser l'organisation des entreprises en groupe. Ce faisant, vous ouvrez la porte aux dérives financières et aux détournements et vous la fermez devant l'obligation d'alerte. en refusant un délai d'application au 1janvier 2022 pour permettre à la profession d'engager sa mutation, vous mettez en péril 3 000 cabinets de proximité et le probable licenciement de 7 000 employés sur tout le territoire français. M. le ministre se gaussait d'une alliance contre nature, selon lui, entre la droite et la gauche sur ces thèmes.

Par ailleurs, le relèvement des seuils pour les entreprises peut s'entendre, sauf que l'occasion est saisie de pénaliser plus encore les salariés et de priver nombre d'entre eux du bénéfice de la participation ou de la protection du règlement intérieur pendant cinq ans au moins, voire, parfois, pour l'éternité. la secrétaire d'État, accorde jusqu'à 50 % des sièges aux salariés dans les conseils d'administration, mais les salariés français n'auront que la portion congrue. congrue. L'élargissement de l'objet de l'entreprise, que l'article 1833 du code civil définit comme servant uniquement l'intérêt commun de ses salariés, est timide : vous avez refusé que les salariés soient, enfin, admis comme l'une des deux parties constituantes. M. le ministre n'est pas avare de déclarations vertueuses sur l'éventail des salaires sur les avantages des dirigeants, dont Tom Enders illustre le caractère inacceptable. Ces condamnations paraîtraient plus sincères s'il n'avait rejeté nos propositions de plafonnement des hauts salaires, de limitation des retraites chapeau et autres stock-options, d'interdiction de versement de dividendes financés par l'emprunt ou à la suite de licenciements. Il est vrai que, en chemin, le Gouvernement a trouvé plus ultra que lui en matière de libéralisme. La majorité de droite n'y était pas allée de main morte relèvement du seuil de cinquante à cent salariés, avec une véritable régression sociale ; refus de toucher à l'objet de l'entreprise sous prétexte de fragilité juridique, argument curieux qui permet d'en rester à la mouture de 1804, remaniée en 1974 une économie sociale brimée par une augmentation de 20 % des cotisations, alors que celles de l'économie conventionnelle seraient divisées par deux. Ce gouvernement affirme souvent : « C'est sans précédent ! C'est rarement une réalité, mais le fait de puiser sans vergogne, à larges mains dans les caisses de la sécurité sociale est, de fait, sans précédent : 500 millions d'euros par la suppression du forfait social,

sur certains éléments. Monsieur Canevet, je vous rassure, il est tout à fait possible de conclure des accords d'intéressement tout au long de l'année : si vous concluez un, par exemple, au troisième trimestre, celui-ci sera applicable pour l'ensemble du deuxième semestre.

Je me réjouis de votre soutien sur les responsabilités sociales de l'entreprise. Je regrette que vous ne mentionniez pas les progrès qu'apporte ce texte sur la parité, la participation des salariés, l'intéressement, la participation des salariés au conseil d'administration,

connivence ». Ce genre d'expression, permettez-moi d'être un peu solennelle, est irresponsable, voire inacceptable, quand bien même elle est censée faire impression sur le peuple. peuple. Ce genre de formules toutes faites, qui font plaisir à tout le monde, explique ce qui se passe aujourd'hui sur les ronds-points ! Pour ma part, je ne me permettrais pas de rebondir sur les revendications des « gilets jaunes » qui souhaitent supprimer cette assemblée, parce que je ne trouve pas que cette revendication soit raisonnable

Hugonet, je me reconnais parfaitement dans la citation du général de Gaulle. Je note d'ailleurs qu'il avait inventé avant tout le monde le « en même temps » : voilà qui me réjouit

mes chers collègues, pour défendre la motion que notre commission spéciale a adoptée sur l'initiative de ses trois rapporteurs, je développerai trois axes : premièrement, la plus-value apportée par le Sénat à l'occasion de l'examen de ce texte, plus-value dont nous pouvons être fiers collectivement ; la situation de blocage qui résulte du texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale ; troisièmement, et enfin, les perspectives, les enseignements que nous pouvons tirer de ce parcours législatif. Commençons par ce qui reste du travail sénatorial sur ce projet de loi. Tout n'est pas négatif dans ce texte. Le Sénat, comme toujours, s'est attaché à produire un travail de qualité. Il a pu « engranger », si j'ose dire, quelques avancées sur chacune des parties du projet de loi, mais trop souvent sur des aspects que je qualifierai de « secondaires Mes collègues rapporteurs Élisabeth Lamure et Michel Canevet ont souligné ces points de satisfaction : ils concernent la dématérialisation des factures d'électricité et de gaz, les tarifs réglementés, les rattrapages de la loi Égalim s'agissant des plastiques et des produits phytopharmaceutiques, l'ouverture en soirée des commerces de détail alimentaires, ou le droit des entreprises en difficulté. Pour ma part, j'évoquerai plusieurs modifications apportées par le Sénat sur la création des reçus d'entreposage, la réforme de l'assurance vie, les crypto-actifs, la réforme du PEA et du PEA-PME, la fiscalité des jeux, la finance solidaire, ou encore l'émission d'actions de préférence. Je crois aussi que nous pouvons nous satisfaire d'avoir introduit des garde-fous et un cadre de régulation pour Aéroports de Paris.

Venons-en à la situation de blocage consécutive au vote de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Celle-ci, de son propre fait ou sur l'initiative du Gouvernement, a détricoté avec méthode quasiment tout ce que le Sénat avait fait en première lecture sur les sujets les plus importants.

c'est plus regrettable lorsque le texte voté par le Sénat en première lecture était un texte de compromis, favorisant l'acceptabilité des dispositions proposées par le Gouvernement dans son projet initial. Or ces cas de figure

tout en conservant les obligations en matière d'institutions représentatives du personnel. Mais rien n'a suivi et cette proposition est restée lettre morte. Quel dommage, madame la secrétaire d'État ! Dans cette situation, il est inutile de reprendre aujourd'hui un débat dont tout le monde a compris qu'il n'aboutirait pas. À ce stade de la navette, après engagement de la procédure accélérée, je le rappelle, nous n'obtiendrons aucune concession supplémentaire de l'Assemblée nationale. Il vaut bien mieux marquer clairement notre désaccord et éviter que la voix de notre assemblée se perde dans la répétition des mêmes arguments. Pour autant, après ce vote, il reste beaucoup à faire. Tout d'abord pour les entreprises, auxquelles ce projet de loi était destiné, puisqu'il était question de favoriser leur croissance et leur transformation. vue, nous ne sommes pas au rendez-vous de l'ambition, et ce texte suscitera sans doute autant de déceptions qu'il a suscité d'espoirs. Qu'il s'agisse des seuils, de la participation et de l'intéressement, de la simplification des procédures, de la compétitivité, ce projet de loi manque incontestablement de souffle. Et je fais devant vous le pari que certaines mesures fortes adoptées par le Sénat finiront par prospérer dans les années à venir. ! Il reste aussi beaucoup à faire en direction de l'opinion et de nos concitoyens. Sur les mesures les plus importantes de ce texte, et malgré ce que l'on nous a présenté comme une concertation exemplaire de plus d'un an, c'est finalement le débat au Sénat en première lecture qui a été le révélateur. Qui parlait de la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des jeux avant que le Sénat ne pose à la fois la question de son contenu, de son bien-fondé et surtout celle de la régulation ?

celui du financement des aides à l'innovation. La vraie raison, c'est la volonté du Gouvernement de contenir la progression de la dette publique et d'obtenir, si possible, sa diminution d'ici la fin du quinquennat. C'est peu de dire qu'il existe une profonde frustration de l'opinion et des sénateurs face à ce débat tronqué. C'est particulièrement dommage dans le contexte actuel de grand débat, sur fond de revendications pour une démocratie plus active.

Nos collègues ont évoqué les lacunes du brouillon de cahier des charges d'ADP. Je prendrai deux autres exemples. Celui des ordonnances, tout d'abord. Il y a dans ce texte, comme dans d'autres, beaucoup trop de demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance.

Mais, pour le reste, j'ai dénombré pas moins de onze habilitations et vingt-sept ratifications dans le texte ! Or, je le rappelle, les ordonnances sont l'instrument par lequel l'exécutif préempte les sujets qui ne seront pas évoqués au Parlement. Les déclarations sur la coconstruction des ordonnances avec les parlementaires sont parfaitement illusoires, madame la secrétaire d'État. Elles ne remplacent aucunement le débat parlementaire, surtout quand la ratification se fait par voie d'amendement. Et elles ne permettent pas non plus d'échanger avec l'Assemblée nationale.

au Gouvernement. Or, à ce jour, tant le périmètre des droits exclusifs confiés à l'opérateur que les contours de la régulation du secteur demeurent incertains. Je continue de penser que rien ne nous assure aujourd'hui que le Gouvernement ne favorisera pas la valorisation de l'entreprise, au détriment des impératifs de santé publique et d'addiction au jeu. Mes chers collègues, compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission spéciale vous invite à voter la motion tendant à opposer la question préalable au présent projet de loi. Pour autant, il nous semble que le Sénat aura une nouvelle fois démontré sa capacité à être un législateur minutieux, précis et vigilant au service de la qualité de la loi. Je veux ici réaffirmer avec force l'utilité et l'intérêt du bicamérisme pour une démocratie vivante et forte, dont la France peut et doit s'enorgueillir !

ne permettrait pas « d'aller plus loin dans la recherche de compromis et de dispositifs plus équilibrés entre les deux assemblées sur les différents volets du texte

Madame, messieurs les rapporteurs, dans l'exposé des motifs de votre motion, vous expliquez que le projet de loi « devait favoriser la croissance et la transformation des entreprises ». L'utilisation de l'imparfait traduit

Cette loi facilitera l'accès des entreprises à des financements diversifiés. Cette loi aidera les entrepreneurs à rebondir. Enfin, cette loi est importante sur le plan social avec, par exemple, la protection des conjoints collaborateurs, le développement de l'actionnariat salarié, le développement de l'épargne salariale et la suppression du forfait social dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

! Au lieu de s'en réjouir et de reconnaître que le texte soumis à notre examen est équilibré, les auteurs de la question préalable continuent de faire des privatisations la pomme de discorde entre les deux chambres. Cet argument est d'autant moins recevable qu'il émane de parlementaires qui, en 2017, ont soutenu un candidat à l'élection présidentielle, qui plaidait pour la reprise des privatisations. Cet argument n'a pas non plus de sens au regard des garanties supplémentaires qui ont été apportées en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et le Gouvernement.

des redevances aéroportuaires le statut d'autorité administrative indépendante, dont elle ne dispose pas aujourd'hui. Enfin, le projet de loi prévoit la possibilité, pour les collectivités territoriales, de déléguer à leur exécutif le droit de prendre des participations au capital d'ADP. L'avenir montrera que ces mesures sont fondées et permettront d'aller de l'avant. Non, la privatisation d'ADP ne porte pas atteinte à la souveraineté de l'État Ce dernier conservera ses missions régaliennes, dont la police aux frontières, le contrôle des douanes, l'autorité de la Direction générale de l'aviation civile. Non, il n'y a pas de monopole naturel pour les aéroports franciliens. Non, la privatisation d'ADP ne reproduira pas les mauvaises pratiques de la privatisation de la gestion des autoroutes, qui a été engagée, il y a quelques années, par la droite.

en 2015 par le gouvernement Valls et qui accorde la neutralité fiscale aux concessionnaires d'autoroutes. Non, la privatisation d'ADP ne devrait pas entraîner de hausse des tarifs des redevances, en dehors de ce qui est prévu. Pour ce qui concerne la privatisation de la Française des jeux, le dispositif soumis à notre examen rend inopérantes les critiques exprimées en première lecture par la majorité sénatoriale. des mesures relatives à la réforme de la fiscalité des jeux d'argent et de hasard- au fond, la Française des jeux est essentiellement une machine à générer du « cash fiscal les députés ont précisé l'habilitation du Gouvernement à refondre la régulation du secteur. La qualité d'autorité de supervision sera ainsi attribuée à la future autorité de régulation unique. Il s'agira d'un grand progrès en matière de contrôle du secteur. Par ailleurs, je note avec satisfaction que treize articles additionnels issus des travaux du Sénat figurent parmi les quatre-vingt-dix-neuf articles qui ont déjà été adoptés conformes. Plusieurs d'entre eux concernent la modernisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Je me réjouis également de constater que d'autres dispositions sénatoriales sont quasi conformes,

s'agissant de l'assurance vie. Le dispositif relatif à la transférabilité des contrats sans conséquence fiscale apparaît tout à fait satisfaisant. De plus, grâce au Sénat, les assureurs auront

à opposer la question préalable, déposée au nom de la commission spéciale. Nous regrettons en effet que la majorité sénatoriale refuse de débattre de nouveau d'un texte d'une telle ampleur. Nous rejetons aussi et dénonçons la surdité du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, en particulier sur la question des privatisations. Comme nous l'avons indiqué lors de la première lecture, madame la secrétaire d'État, le modèle économique et social que nous défendons est à l'opposé de votre projet de loi, qui promeut la financiarisation de l'entreprise et de la société, en général. Alors que notre pays aspire à plus de justice, justice fiscale, justice sociale, mais aussi justice au sein de l'entreprise, c'est finalement l'injustice sociale que vous érigez en modèle de réussite au nom d'une certaine conception de la compétitivité Alors que nos concitoyens rejettent en bloc la destruction ordonnée des services publics qui ont fait de notre pays un véritable modèle, vous continuez dans la voie du désengagement de l'État. Vous faites le choix de la dérégulation, au risque de fragiliser l'ensemble de nos PME. Vous prétendez vouloir libérer les entreprises, en particulier les plus petites. Pourtant, rien dans ce texte ne remet en cause la domination des grands groupes donneurs d'ordre, qui pressurent au quotidien nombre de ces nombre de ces entreprises. Rien sur la sous-traitance, rien sur la chaîne de valeur ! Enfin, et c'est le coeur de notre opposition, ce projet de loi accélère le désengagement de l'État, garant d'un certain ordre économique, mais aussi de l'État actionnaire. Il y a de trop nombreux renoncements dans ce texte. Vous renoncez à contrôler les jeux d'argent. Vous renoncez à un service public de l'énergie à l'heure ou la précarité énergétique n'a jamais été aussi forte dans notre pays. Vous renoncez à la véritable maîtrise publique du transport aérien. C'est sans doute pourquoi ce texte ne passe pas. Au milieu d'un grand débat au cours duquel vos orientations ont été sévèrement critiquées, vous faites preuve d'un entêtement d'un aveuglement qui défient toute rationalité et pèsent sur tout choix futur de politiques publiques différentes. La fronde gronde de toute part contre ces privatisations, qui sont un non-sens constitutionnel, économique, stratégique,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

Nous ne souhaitons pas faire de la surenchère et nous ne voulons pas nous soumettre à une telle forme d'instrumentalisation et de récupération.

survient en clôture de l'examen du projet de loi Pacte. Je regrette l'appropriation personnelle, parfois, et médiatique qu'elle suscite. Pour revenir au texte de loi lui-même,